La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire issue des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est tenue au Sénat le 8 janvier dernier. Déjouant les pronostics de nombreux commentateurs, nous sommes parvenus, députés et sénateurs, à un accord unanime sur un texte très attendu par nos concitoyens et que la navette parlementaire a enrichi et équilibré. À mon sens, cet accord exigeant que nous avons trouvé constitue une double bonne nouvelle. Premièrement, il révèle que nous sommes, nous parlementaires, en phase avec une demande sociétale très forte d'un changement radical de notre modèle de production et de consommation, pour en finir avec le « tout-jetable », en donnant à tous les acteurs concernés les outils nécessaires pour accomplir la transition vers un nouveau modèle d'économie circulaire et de lutte contre le gaspillage de nos ressources. le sujet du plastique est emblématique. Sans tomber dans le « plastique-bashing » systématique, nous devons agir vite, guidés par une forte dynamique européenne, afin d'en finir avec les emballages à usage unique et les microplastiques qui polluent les océans. Deuxièmement, cet accord démontre toute la force de notre parlementarisme bicaméral. L'examen de ce projet de loi a donné lieu à une lecture dans chaque assemblée et à l'instauration d'un véritable dialogue. Le Sénat, saisi en premier, a ouvert la voie sur de nombreux sujets et, sur d'autres, a suscité de sains débats. L'Assemblée nationale a apporté des enrichissements et poursuivi notre dynamique.

du texte. Le projet de loi initial, qui ne comportait que treize articles, n'était peut-être pas à la hauteur des enjeux et des attentes des Français. Le travail des deux chambres a permis de lui donner une véritable envergure. Malgré des positions parfois fortement exprimées, nos deux assemblées ont su travailler dans le respect mutuel et dans le souci d'affirmer une véritable ambition environnementale. La navette n'a pas été caricaturale : il n'y a eu ni chambre d'enregistrement du projet gouvernemental ni volonté de détricotage stérile. Avant d'en venir aux dispositions essentielles de ce projet de loi, j'ajoute que ce travail parlementaire a été largement transpartisan. Tous les groupes politiques se sont mobilisés pour enrichir un texte qui comporte aujourd'hui les apports et les solutions de chacun. Je pense à la fin de la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et les locaux à usage professionnel, votée par le Sénat sur l'initiative de nos collègues Sophie Primas et Didier Mandelli ; au plan de lutte contre les microplastiques dans l'environnement, proposé par les élus du groupe socialiste ; aux objectifs ambitieux en matière de prévention et de gestion des déchets, adoptés sur l'initiative de notre collègue Jean-François Husson aux dispositions sur l'obsolescence logicielle émanant du groupe communiste ; au renforcement des objectifs nationaux de valorisation énergétique des déchets non recyclables, l'initiative du groupe centriste ; à l'identification des sites opportuns pour installer des fontaines, en remplacement des bouteilles plastiques, dans les schémas de distribution d'eau potable, grâce à notre collègue du groupe Les Indépendants- République et Territoires, Jérôme Bignon Bignon ; aux dispositions visant à favoriser le don des invendus non alimentaires de première nécessité aux associations de lutte contre la précarité, introduites sur la proposition de notre collègue du RDSE, Ronan Dantec. Cette énumération n'est pas anecdotique. Elle reflète un véritable travail, construit sur toutes les travées de notre hémicycle, et qui demeure dans le texte définitif. Concernant le fond du texte, j'insisterai sur trois points. En premier lieu, nous sommes parvenus, me semble-t-il, à un texte plus ambitieux, et surtout plus transversal, que le projet de loi initial : l'économie circulaire doit irriguer toutes nos politiques publiques. Initialement composé de treize articles dédiés à l'information du consommateur, à la lutte contre le gaspillage non alimentaire et à la responsabilité des producteurs, le projet de loi a vu son champ considérablement élargi sur l'initiative du Sénat.

-, des objectifs en termes de prévention et de gestion des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore de l'exemplarité de l'État la commande publique. Sénat a adopté la création de deux fonds importants : un fonds dédié à la réparation et un fonds pour le réemploi solidaire. Nous avons également renforcé les droits et l'information du consommateur, avec, par exemple, la création d'un indice de durabilité, complété par l'Assemblée nationale. En deuxième lieu, notre travail a permis l'adoption d'un texte plus équilibré. En témoigne le traitement de la question des déchets du bâtiment, sujet en réalité indissociable de la lutte contre les dépôts sauvages : nous avons abouti à un système garantissant une responsabilité

l'établissement d'un maillage territorial de points de reprise soit rendu obligatoire pour la filière, ainsi qu'une contribution des producteurs à l'ouverture de nouveaux points de collecte et à l'extension des horaires des points de collecte existants. Sur le sujet de discussion le plus sensible entre les deux assemblées, à savoir la consigne pour recyclage, nous sommes également parvenus à un équilibre qui permettra aux collectivités territoriales d'achever le déploiement de l'extension des consignes de tri avant de devoir justifier de leur capacité à atteindre les objectifs européens en matière de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique sans mettre en place de dispositif de consigne. En la matière, le Sénat a joué un rôle essentiel : il a veillé à ce que le service public de gestion des déchets ne soit ni désorganisé, ni affaibli, ni remis en cause par un dispositif dont la plus-value environnementale paraît limitée. Nous avons relayé les inquiétudes légitimes des collectivités territoriales, qui assument cette mission avec beaucoup d'efficacité depuis de nombreuses années et ont massivement investi afin d'être aussi performantes que possible. possible. Toutefois, tout le monde devra jouer le jeu. Le dialogue devra se poursuivre avec les collectivités territoriales et les moyens devront être effectivement mis à leur disposition afin qu'elles puissent atteindre les objectifs fixés. Nous y veillerons : nous le devons. dernier lieu, cet accord est exigeant. Des objectifs ont été fixés. Beaucoup de mesures devront trouver à s'appliquer par le biais de dispositions réglementaires. Je souhaite que le Sénat puisse veiller au suivi de l'application de toutes ces mesures et que le Gouvernement s'engage à nous associer à cet indispensable travail d'évaluation : nous y serons attentifs ! La parole est

C'est le moins que l'on puisse dire ! Certes, mais justement, grâce à nos désaccords, malgré nos positions parfois éloignées, malgré des invectives inutiles, je suis fière de ce texte anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont, ensemble, nous avons révélé tout le

Le texte sur lequel vous vous prononcerez dans quelques minutes a vu sa taille multipliée par dix, en grande partie grâce à vos ajouts. Ce texte, vous et moi pouvons en être fiers.

Ce fléau, nous l'endiguerons grâce aux dispositions que vous avez introduites, comme l'attribution de nouveaux moyens de police et de répression aux maires et aux présidents d'intercommunalité. Nous l'endiguerons aussi grâce à la mise en place de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits du bâtiment. C'est un levier indispensable de financement de la reprise gratuite des déchets triés

le potentiel des outils et technologies dont elles disposent aujourd'hui- l'extension des consignes de tri -, et, dans un second temps, nous procéderons à une analyse objective de la situation. Cette analyse pourrait conduire à la mise en oeuvre d'un dispositif de consigne qui soit un accélérateur de la transition

À cette occasion, j'avais affirmé mes réserves concernant ces mesures : j'approuvais les objectifs, mais doutais des moyens. Comme vous avez pu le constater, nous ne les avons pas abandonnées. Elles ont été

l'Assemblée nationale et du Sénat. Ainsi, nous avons pris des mesures fortes au sujet des perturbateurs endocriniens, pour rendre leur présence dans la composition des produits entièrement transparente. Nous avons mis en place une stratégie de sortie du plastique à usage unique en vingt ans,

dès le 31 décembre 2024. Quelle audace ! Ce projet de loi consacre notre volonté collective de construire une écologie du quotidien, une écologie du rassemblement, qui ouvre la porte à des transformations systémiques tout en valorisant chaque geste

Aujourd'hui, l'économie mondiale n'est que circulaire de 8,6 %. Il y a tout juste deux ans, elle l'était de 9,1 %. L'écart mondial de circularité se creuse. Il y a des raisons à cette tendance négative, mais le résultat reste le même : les nouvelles ne sont pas seulement mauvaises, elles sont pires. La tendance négative globale peut s'expliquer par plusieurs tendances profondément ancrées dans la tradition de l'économie linéaire, qui consiste à " créer des déchets ". Nous avons désespérément besoin de solutions transformatrices et correctrices ; le changement est une obligation. Ce changement, c'est celui qui s'incarne au travers du texte que nous allons voter aujourd'hui. Il traduit la volonté de prévenir une dégradation environnementale accélérée tout en luttant contre les inégalités sociales. L'objectif final est de créer un espace opérationnel écologiquement sûr et socialement juste pour nos concitoyens. Comme le prévoient les objectifs de développement durable et l'accord de Paris, les pays ont un rôle pivot à jouer. Madame la secrétaire d'État, ce texte nous permettra d'accélérer le changement de notre modèle de production et de consommation afin de réduire le volume de nos déchets et de préserver notre environnement. Après les lectures successives au Sénat et à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire s'est réunie le 8 janvier dernier. Elle est parvenue à un accord adopté à l'unanimité. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec nos collègues députés. Je salue en particulier les efforts de notre rapporteure, Marta de Cidrac,

Le texte auquel nous sommes parvenus me semble parfaitement équilibré. Nous avons conservé les dispositions essentielles adoptées par l'une et l'autre chambres, notamment nombre d'avancées défendues par la Haute Assemblée. Je le

premier impératif est de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne. Les mesures que nous avons adoptées pour l'information des consommateurs vont dans ce sens, avec des obligations d'étiquetage et la création de nouveaux indices de réparabilité et de durabilité, qui auront des répercussions dans notre vie quotidienne : les consommateurs seront éclairés quant aux conséquences de leurs choix, et ce premier pas a toute

Nous avons également engagé un combat contre le gaspillage indécent de ressources que constitue l'utilisation du plastique à usage unique et accru les possibilités et les obligations en matière de recours au réemploi, par toute une série d'objectifs et de mesures concrètes. Nous avons renforcé la lutte contre le gaspillage alimentaire et adopté des mesures pour mettre un terme à la pratique scandaleuse de la destruction des invendus non alimentaires. La commission mixte paritaire a confirmé le renforcement du pouvoir des maires et des collectivités territoriales pour lutter contre les dépôts sauvages. Enfin, s'agissant du tri et de la consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, qui ont suscité tant de débats passionnés, pour ne pas dire plus, la commission mixte paritaire est parvenue, me semble-t-il, à un accord équilibré. La voie médiane trouvée avec nos collègues députés devrait permettre d'atteindre nos objectifs de recyclage tout en respectant les demandes des collectivités territoriales, qui avaient, plus que légitimement, exprimé des inquiétudes. Elles ont été entendues, et je me réjouis que cette solution, plaçant les collectivités au coeur du dispositif, ait été trouvée.

avec ce texte, notre pays se dote d'une boîte à outils qui doit lui permettre d'avancer à marche forcée, partagée et raisonnée vers une transition écologique que nous appelons tous de nos voeux et des modèles de consommation plus vertueux. Le texte voté, il importera d'en déployer sans tarder les avancées et les mesures sur tout le territoire national, pour une véritable mobilisation générale des comportements. À cet égard, mettre en oeuvre, à l'instar de la démarche France Mobilités,

Nous disposons d'un savoir-faire, mais le faire-savoir est essentiel pour partager toujours davantage la nécessaire transition écologique. Lutter contre le gaspillage et pour une économie circulaire : voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Vous pouvez compter sur l'engagement du groupe La République En Marche pour relever à vos côtés ce beau défi, madame la secrétaire

Par ailleurs, dans sa grande sagesse, le Sénat a rejeté la consigne pour recyclage plastique, qui suscitait l'indignation légitime des acteurs du secteur. Il faut le dire, cette mesure reflétait la puissance des lobbies qui, avec votre complicité,

Je pense à la lutte contre l'obsolescence programmée, et notamment logicielle, à la définition du vrac et à sa promotion, à la lutte contre le suremballage et le gaspillage des invendus par la création d'un fonds de réemploi, même si la portée de cet outil a été fortement limitée. Je pense également à la promotion

qui souffrent d'exposition à des matières nocives pour la santé. Deux sujets ont particulièrement polarisé nos débats : la lutte contre le plastique et la consigne. Le Sénat avait adopté notre amendement tendant à rétablir la véritable consigne, c'est-à-dire celle du verre dans les cafés, hôtels et restaurants, qui prévalait jusqu'en 1989. La seconde délibération est

sujet du plastique, les débats ont permis de sortir de la seule problématique du recyclage, pour aller vers une interdiction pure et simple. Nous sommes satisfaits d'avoir pu élargir les termes du débat en passant d'une discussion sur les contenants,

était nécessaire pour protéger notre environnement et lutter contre la pollution, due notamment à nos déchets. Nous ne cessons de le rappeler depuis des mois, et je le redis avec force en ce mois de janvier 2020 : les prévisions pour 2050 en matière de réchauffement climatique

Nous resterons toutefois attentifs aux évolutions et aux effets attendus. Le groupe Les Indépendants a, dès le début des discussions, mis en avant l'enjeu primordial du régime de la responsabilité élargie du producteur.

le compromis trouvé nous semble équilibré. Les collectivités territoriales ayant mis en place des dispositifs spécifiques auront la possibilité de produire des résultats et d'amortir leurs investissements. Si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints, des consignes de bouteilles plastiques seront mises en place en 2023. Dans mon département, la Seine-et-Marne, de nombreuses collectivités territoriales ont investi et le système fonctionne très bien

la réduction du gaspillage des médicaments et du gaspillage alimentaire, la promotion du réemploi et de la réparabilité ou encore l'information des consommateurs, clé de la compréhension et des choix éclairés nous devons donc poursuivre les efforts en ce sens. Nous saluons également les dispositions prises afin d'aider les communes à lutter contre les dépôts sauvages. Il s'agit d'un point important pour nos territoires et pour nos maires.

Comme nous avons pu le dire, chacun d'entre nous est concerné par les évolutions et les efforts à mettre en oeuvre. L'État, les industriels et les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, doivent contribuer à la circularité de notre économie. Notre vigilance et nos comportements nous engagent pour la protection de notre environnement, qui, comme nous le voyons chaque jour, se détériore. Il reste encore tant à faire Le groupe Les Indépendants votera ce texte, mais nous gardons à l'esprit que la pose de cette première pierre de l'édifice de l'économie circulaire nous oblige à bâtir un dispositif plus vaste dont l'efficacité doit être certaine. Il y va de notre futur !

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous concluons aujourd'hui le parcours législatif d'un texte attendu et nécessaire. L'économie circulaire, jusqu'alors abordée par petites touches dans différents textes, fait enfin l'objet d'une loi spécifique. De nombreuses mesures vont dans le bon sens, en matière d'information du consommateur, d'interdiction de l'élimination des invendus, de réparabilité, de disponibilité des pièces détachées, d'élargissement des REP, de reprise des produits usagés ou encore d'éco-modulation. C'est pourquoi la majorité du groupe Union Centriste votera en faveur de l'adoption de ce texte. Des défis demeurent toutefois devant nous, notamment en matière de prévention des déchets. Le meilleur des déchets, nous le savons, c'est celui qu'on ne produit pas

défis en matière d'optimisation de la collecte, de tri et de recyclage de tous les déchets. Dans cette perspective, quel meilleur outil que les services publics de gestion globale des déchets qui existent sur tous les territoires ? Vous le savez, madame la secrétaire d'État, aux yeux d'une majorité de sénateurs et d'élus des collectivités locales, la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est une mesure à double tranchant c'est d'ailleurs pourquoi ce sujet a pris une place aussi importante dans nos débats. Sous prétexte de permettre la collecte de 90 % des bouteilles en plastique d'ici à 2029, elle conduit à cautionner, de fait, la poursuite de l'usage du plastique par les industriels de la boisson pendant les dix années à venir, elle met à la charge du consommateur un coût supplémentaire, elle induit une démultiplication des circuits de collecte, techniquement et financièrement, les services publics existants qui assurent la gestion de tous les déchets. Certes, nous l'avons dit, le système actuel de collecte doit être amélioré, mais il est fondé sur un maillage territorial construit et modernisé depuis plus de vingt ans par les collectivités de proximité, qui sont responsables et réactives. Des efforts financiers colossaux ont été consentis pour mutualiser des dispositifs de collecte, de tri et de recyclage permettant la prise en charge de l'ensemble des déchets des ménages sur tous les territoires, à des coûts supportables pour les contribuables locaux. L'extension des consignes de tri en cours de déploiement et le tri cinq flux hors foyer, à ce jour insuffisamment répandu dans les commerces et les entreprises, doivent faciliter la collecte dans les années à venir et permettre d'améliorer les performances, déjà proches de 90 % dans certains territoires innovants. Enfin, pour développer les dispositifs de proximité existants, mutualisés, économes et efficaces, économiquement comme écologiquement, nous comptons sur votre vigilance, madame la secrétaire d'État, à l'égard de la gouvernance des éco-organismes, et singulièrement de Citeo, qui doit renforcer la collégialité en son sein pour créer un climat de confiance et soutenir davantage les collectivités.

la tournure qu'ont prise les débats et a permis de placer la focale sur les territoires et les collectivités chargées de la gestion des déchets. Je veux bien sûr parler de l'affaire de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, qui a constitué l'une des pommes de discorde et a monopolisé le débat. Cette mesure, inspirée par les grands industriels de la boisson, aura tout de même permis au Sénat de faire de la lutte contre les emballages en plastique l'un des axes structurants de ce projet de loi, initialement muet sur ce point.

2030 que nous avions fixés. Désormais, le texte indique simplement que « la France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040 ». ne donne pas un cadre clair aux industriels et semble déjà excuser un futur échec ! Alors que la discussion de ce texte a eu le mérite de sensibiliser nos concitoyens et d'interroger nos modes de consommation et que les initiatives locales se multiplient dans nos territoires, il est dommage de ne pas capitaliser sur cet engouement populaire dans la loi.

cela aurait laissé à la majorité de l'Assemblée nationale et au Gouvernement les mains libres pour aller à l'encontre de la volonté des collectivités territoriales. À ce propos, madame la secrétaire d'État, je tiens à préciser que les associations représentant celles-ci ne sont pas des lobbies. Très bien ! Cette tentative de disqualification auprès de l'opinion publique a beaucoup ému dans les territoires.

d'utilisation de ressources renouvelables, de recyclabilité ou de présence de substances dangereuses. Des manques importants subsistent. Je pense au compteur d'usage pour les appareils électroménagers, dont nous avions réussi à faire adopter ici ou à l'interdiction des plastiques fabriqués à partir de substances contenant des perturbateurs endocriniens avérés. Néanmoins, l'information du consommateur à ce sujet, notamment des femmes enceintes, progressera grâce à ce texte. Autre point essentiel, la lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire fait un bond en avant, avec l'interdiction, au titre II, de détruire les invendus,

Par ailleurs, le fonds national unique de réemploi solidaire, dont nous avions voté des deux mains la création, a été supprimé, au profit d'un dispositif à la main des éco-organismes, et donc des producteurs. C'est dommage pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui attendait un signal de confiance dans le domaine de la lutte contre les dépôts sauvages, nous pouvons saluer la mise en place de nouveaux outils efficaces qui faciliteront le combat quotidien des élus locaux contre ce véritable fléau. Même s'il manque un volet éducatif et pédagogique, nous avons abouti à un texte plus équilibré, tout compte fait favorable à la montée progressive d'une économie à tout le moins plus circulaire, sans qu'il s'agisse pour autant du grand tournant écologique qu'attendent les Français, qui y sont prêts.

Lors de la lecture au Sénat, j'avais émis des doutes sur la rédaction issue de nos débats, qui selon moi laissait toute latitude aux industriels pour mettre en place une consigne pour recyclage sans aucun encadrement. Le compromis trouvé laisse finalement aux collectivités territoriales et aux recycleurs jusqu'à 2023 pour tenter d'atteindre les objectifs de collecte, la CMP considérant que des efforts ont déjà été entrepris et qu'il serait préjudiciable pour tous de s'engager dans une autre voie avant une première évaluation. Néanmoins, compte tenu de l'urgence, un dispositif de consigne pourrait être mis en place après 2023 si le bilan des performances de collecte n'était pas satisfaisant. Il s'agit bien d'un compromis, car il s'inscrit dans le respect des engagements et des investissements consentis par les collectivités, tout en rappelant que l'objectif final, à savoir recycler 100 % de nos déchets plastiques d'ici à 2025, Sur ce même sujet, il paraît indispensable d'optimiser la collecte des déchets produits hors foyer, qui demeure, dans notre pays, largement en deçà des ambitions européennes. Ayant défendu un amendement en ce sens, nous nous réjouissons de l'inscription dans le texte de la généralisation de la collecte séparée des déchets produits hors foyer d'ici à 2025. qui concerne les dépôts sauvages, de nettes améliorations sont prévues, notamment le renforcement des pouvoirs de police du maire, la création d'une amende forfaitaire de 1 500 euros dont le produit reviendra aux communes,

Ces mesures nous permettent de saluer les efforts des maires dans ce domaine et de les conforter dans leur rôle, tout en les protégeant davantage afin que le drame survenu l'été dernier à Signes ne puisse se reproduire. S'agissant de l'engagement des collectivités territoriales et des administrations dans l'économie circulaire, nous saluons les objectifs de réduction de la consommation de plastiques à usage unique et de la production de déchets, ainsi que la valorisation des biens issus de l'économie circulaire. Ainsi, à compter de 2021, au moins 20 % des biens acquis annuellement par les services de l'État ou par les collectivités territoriales devront être issus du réemploi ou intégrer des matières recyclées. La commande publique devra prendre en compte le recours à des matériaux issus du réemploi et la priorité sera donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés lors du renouvellement des flottes de véhicules, une mesure que j'avais défendue avec mon collègue Didier Mandelli.

interdisant, dès 2023, l'impression des tickets papier lors d'un achat, restreignant la consommation d'eau potable dans les bâtiments neufs ou encore prohibant la mise sur le marché de toute substance en l'état de microplastiques, dont on sait qu'ils font beaucoup de dégâts, notamment lorsqu'ils sont ingérés par la faune aquatique. en mettant en exergue les mesures permettant au consommateur de s'orienter vers des produits écologiquement plus vertueux, par l'amélioration des consignes de tri et de l'information du client sur les qualités environnementales des produits et leur indice de réparabilité, la mise à disposition de pièces détachées plus rapidement et plus longtemps ou l'incitation à recourir à des contenants réutilisables. Nous savons en effet que c'est le consommateur qui guide les principales évolutions du secteur industriel et qui engage toute la société à s'inscrire dans une démarche vertueuse, celle de l'économie circulaire.

Les objectifs sont également affichés clairement, avec des dates butoirs qui nous engagent. Ce texte ne doit toutefois pas nous faire oublier l'urgence climatique, les niveaux de pollution de notre planète et la nécessité de faire évoluer notre mode de vie. La parole

Après une longue et riche période de concertation et la mise en place d'un comité de pilotage, auquel j'ai pu participer en tant que président du groupe d'études sur l'économie circulaire du Sénat, l'examen de ce projet de loi, qui marque une avancée majeure sur le sujet, arrive enfin à son terme. La première mouture de ce texte, qui comportait six articles et deux ordonnances intégrant les principales mesures, nous avait conduits, Hervé Maurey et moi-même, à réagir pour demander la tenue d'un débat plus conforme aux attentes légitimes du Parlement. Nous avons sans doute eu raison de le faire, si l'on en juge par l'enrichissement du texte, passé de 13 articles initialement à 87 après son adoption par le Sénat puis à 131 après son examen à l'Assemblée nationale.

Nous partagions toutefois les mêmes objectifs, nos différences d'appréciation portant sur les moyens à engager et le rythme de leur mise en oeuvre. Notre rapporteure, Marta de Cidrac, a parfaitement rempli sa mission en auditionnant la quasi-totalité des acteurs concernés, en prenant la pleine mesure des enjeux de ce texte et en présentant à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, puis à nos collègues en séance publique, une vision empreinte de pragmatisme et d'ambition ; qu'elle

De même que le mot « écologie » ne figurait pas dans le dictionnaire en 1974, quand René Dumont s'est présenté à l'élection présidentielle, la notion d'économie circulaire, que je promeus à titre personnel sur les plans professionnel et politique depuis près de trente ans, n'était pas encore entrée dans le champ lexical c'est aujourd'hui chose faite. Il s'agit non pas d'un concept, mais d'une réalité, qui n'est en fait que l'expression de ce que l'on appelle le bon sens et qui apparaît comme une évidence. C'est la traduction du principe « penser global, agir local » et l'essence même du développement durable, conciliant respect de l'environnement, développement économique et approche sociale.

Il se conjugue à toutes les démarches engagées, pour certaines depuis longtemps, par nos concitoyens, les associations, les entreprises et les collectivités. Le chemin est encore long pour parvenir à l'équilibre parfait qui permettrait aux 8 milliards d'habitants de la planète de vivre et de s'épanouir dans de bonnes conditions sans épuiser les ressources naturelles.

dont le Sénat a été un important pourvoyeur n'a pas été sacrifiée sur l'autel du sujet polémique de la consigne : la commission mixte paritaire est ainsi parvenue à dégager un compromis, le 8 janvier dernier.

renforcer l'information du consommateur, la prévention des déchets, la réduction des emballages à usage unique, la lutte contre le gaspillage ou le développement du réemploi et de la réparation,

cet enjeu majeur pour notre société, vous avez fait montre, madame la secrétaire d'État, de volontarisme. Les deux assemblées s'étant déjà accordées sur de nombreux points, la commission mixte paritaire avait pour objet principal de trouver un accord sur la consigne pour les bouteilles en plastique, sujet de blocage entre nos deux chambres. Si le Sénat, avec plusieurs associations environnementales, était réservé sur l'introduction de cette consigne pour recyclage, c'était de crainte que cette dernière ne conduise à une augmentation de la consommation de plastique, nous maintenant ainsi dans l'ère du « tout-jetable

En effet, ces dernières ont investi dans des centres de tri des bouteilles en plastique et revendent les bouteilles collectées dans ces centres à des recycleurs ; la mise en place de la consigne de recyclage signifierait pour elles la perte de ces revenus. Toutefois,

Outre les avancées réalisées en matière de consigne, il faut se féliciter également de l'extension de la responsabilité élargie des producteurs aux produits et matériaux du bâtiment, ainsi que de la reprise gratuite de l'ensemble de ces produits et matériaux.

mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne ne demande la parole ?